de la loi relative à l'extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse, d'autre part, de la loi relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle.

Le 22 août 2009, lors d'une colonie de vacances aux États-Unis, deux jeunes filles, Léa et Orane, ont perdu la vie dans un accident de la route. Cet accident a donné lieu à un rapport de l'inspection générale de la jeunesse et des sports, qui a établi un certain nombre de préconisations,

de mineurs organisé aux États-Unis a donné lieu, outre des enquêtes et procédures administratives et judiciaires, à un rapport de l'inspection générale de la jeunesse et des sports, remis en décembre 2013. Dans ce rapport, un certain nombre de préconisations sont formulées visant à améliorer la sécurité des mineurs, notamment la création, pour les séjours itinérants de mineurs se déroulant à l'étranger, d'un régime de déclaration renforcée fondé sur des critères essentiels, éventuellement issus d'une charte. Je veux vous assurer que la protection des mineurs en accueil collectif à caractère éducatif, dont font partie les séjours de vacances à l'étranger, est une priorité pour le Gouvernement. Les organisateurs de ces séjours sont déjà soumis à une obligation de déclaration de leur accueil, ce qui permet aux services de l'État de vérifier le respect de la réglementation. Cette déclaration comprend des informations relatives à l'organisateur, aux modalités d'accueil, au public accueilli ainsi qu'aux personnes qui assurent l'encadrement des mineurs. Elle comprend également des précisions s'agissant de la date et du lieu des étapes lorsque le séjour est itinérant. Dans le cas d'un séjour à l'étranger, les représentations françaises dans les pays concernés sont systématiquement informées des conditions dans lesquelles ces séjours vont se dérouler. Par ailleurs, afin d'améliorer encore la sécurité des mineurs des mineurs participant à des séjours de vacances à l'étranger, de nouvelles mesures ont d'ores et déjà été prises ou sont en passe de l'être. À titre d'exemple, la réglementation prévoit depuis 2015 que toutes les sessions de formation au BAFA-BAFD- le brevet peuvent être organisées à l'étranger. Ces sessions permettent de mieux appréhender les enjeux et les spécificités des séjours de vacances à l'étranger. Un renforcement des conditions de déclaration est également à l'étude avec les organisateurs de ce type de séjours. Il pourrait par exemple s'agir d'imposer l'obligation de fournir des informations précises sur les modalités de transport mises en oeuvre. Enfin, depuis le 15 janvier dernier, l'autorisation de sortie du territoire pour les mineurs quittant le territoire national sans être accompagnés d'un titulaire de l'autorité parentale a été établie, ce qui renforce également leur

l'avion pour venir à Paris. La question s'adresse à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, et porte sur la nécessité de rendre pleinement applicable, sur le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article R. 123-20 du code de l'organisation judiciaire, les termes : « Il est institué auprès de chaque greffe, pour les opérations dont celui-ci est chargé autres que celles mentionnées à la section 2 une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics Afin de soutenir l'activité du secteur du bâtiment et des travaux publics à Wallis-et-Futuna, il est apparu indispensable de mettre en place une régie pour le recouvrement des créances par voie de saisie-arrêt des rémunérations, afin de réactiver le dispositif du Fonds de garantie à l'habitat. En 2014, le Gouvernement a donc instauré une sous-régie auprès du tribunal de Mata Utu, celle-ci étant rattachée au tribunal de première instance de Nouméa. Or il s'avère que cette solution présente des inconvénients majeurs du fait de l'éloignement des sites. Il conviendrait par conséquent de créer une véritable régie auprès du greffe du tribunal de première instance de Mata Utu, conformément à ce que prévoit l'article R. 123-20 du code de l'organisation judiciaire. Nous

pour mettre en oeuvre le recouvrement des créances par la saisie des rémunérations, préalable nécessaire à la mise en place des prêts à l'habitat. Le code de l'organisation judiciaire prévoit bien qu'il est institué auprès de chaque greffe une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics. Cependant, cette disposition n'est pas applicable à Wallis-et-Futuna, compte tenu des dispositions d'adaptation prévues à l'article R. 531-1 de ce code. La création d'une La création d'une régie supposait donc une réforme profonde par un décret en Conseil d'État. Pour éviter cette procédure, les directions des finances publiques de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, relayées par la cour d'appel de Nouméa, ont invité le ministère de la justice à instaurer, par arrêté, une sous-régie à Mata Utu, rattachée au tribunal de première instance de Nouméa. Mais la fragilité juridique inhérente à une sous-régie ainsi que l'incompatibilité des logiciels utilisés par le régisseur de Nouméa et par la sous-régie de Mata Utu représentaient des obstacles juridiques et techniques au bon fonctionnement de cette dernière. Les chefs de la cour d'appel de Nouméa ont en conséquence demandé la création d'une régie à part entière à Mata Utu en 2015. La Chancellerie a répondu favorablement à cette demande, avec pour objectif une ouverture de la régie dans le courant du premier semestre 2017. Un projet de décret en Conseil d'État d'État est en cours de rédaction au sein des services de la Chancellerie, décret qui intégrera une modification de l'article R. 531-1. Les ministères des finances et des outre-mer ont été saisis de ce projet de réforme. Les chefs de la cour d'appel de Nouméa sont par ailleurs étroitement informés de ce projet,

un demi-siècle, les Chagossiens n'ont jamais cessé de revendiquer leur droit intangible de retourner vivre aux Chagos. Après avoir procédé, en 1965, à l'excision de l'archipel des Chagos du territoire de Maurice, encore colonie britannique, la Grande-Bretagne a cédé, au moyen d'un l'île de Diego Garcia aux États-Unis pour une durée initiale de cinquante ans, reconductible par périodes de vingt ans. Les Chagossiens ont été abandonnés, déracinés et ont vécu misérablement dans des bidonvilles.

de la Chambre des Lords. L'année 2016, cruciale, était celle du renouvellement du bail de Diego Garcia. Le gouvernement de Londres avait laissé nourrir l'espoir d'un avenant au bail permettant une réinstallation maîtrisée des Chagossiens aux Chagos. Il avait même commandé une étude de faisabilité sur les conditions du retour, qui avait conclu positivement. Par ailleurs, Mme Theresa May s'était engagée en octobre 2016, à la veille de l'assemblée générale de l'ONU, à ouvrir la négociation avec Maurice et les Chagossiens. Toutefois, au mépris de ces engagements, le 16 novembre dernier, Londres a brutalement opposé un non définitif à la revendication légitime des Chagossiens. Le bail liant la Grande-Bretagne aux États-Unis a été renouvelé que soit saisie l'occasion historique de réparer le crime. Pour autant, la lutte des Chagossiens n'est pas brisée. Ils crient leur révolte et leur souffrance.

Je voudrais tout d'abord apporter quelques précisions sur ce différend qui oppose le Royaume-Uni et la République de Maurice, différend sur lequel le gouvernement français ne saurait prendre position. Le gouvernement mauricien revendique cet archipel de l'océan Indien, dont la population a été déplacée entre 1965 et 1973. Louée par le Royaume-Uni aux États-Unis, Diego Garcia, la principale île des Chagos, est devenue une base militaire américaine. Depuis leur départ forcé, les Chagossiens, estimés à 9 000 personnes, vivent principalement à Maurice, aux Seychelles et au Royaume-Uni. Soyez assurée, madame la sénatrice, que la France n'est pas indifférente au sort des Chagossiens. Après plus de quarante ans d'exil, les Chagossiens et leurs descendants continuent de rencontrer des difficultés d'insertion économique et sociale. Le devenir de cette population déplacée doit, bien sûr, être pris en compte lors de la résolution du différend relatif à la souveraineté des Chagos.

En outre, ma question portant sur l'utilisation abusive et le détournement des textes européens en matière de salariés détachés par certaines compagnies aériennes, une grande partie de la réponse ne pourra être apportée qu'au niveau communautaire. Alors que les compagnies Vueling et Ryanair ont été récemment condamnées par la justice française pour travail dissimulé pour des faits remontant à plusieurs années, la Commission européenne, à la suite de plaintes déposées auprès d'elle par les compagnies concernées, a ouvert une procédure contre la France et lui demande de reconnaître les formulaires de détachement, dits E101 et E102, délivrés par l'Espagne et l'Irlande pour les personnels de Vueling et Ryanair, en application du droit européen. Ce recours aux règles du détachement de salariés par les compagnies aériennes établies dans d'autres pays de l'Union européenne, mais qui opèrent au départ de la France, date d'une quinzaine d'années. Si la pratique du recours à ce statut a d'abord pris la forme d'une prestation de service, elle s'est ensuite transformée en une activité habituelle, stable et continue, et, de fait, contraire au cadre juridique du détachement. En effet, les personnels exerçant en France et prétendument détachés d'Espagne par Vueling et d'Irlande par Ryanair ne résidaient ni en Espagne ni en Irlande, et ne s'y rendaient pas non plus dans le cadre de leurs activités professionnelles. Ainsi, les règles du détachement ont été détournées de leur finalité initiale afin de profiter du système social le plus avantageux. Compte tenu de la situation du pavillon aérien français, il serait souhaitable de renforcer les contrôles par les pouvoirs publics de ces transporteurs pour vérifier l'application des règles sociales françaises et l'absence de recours abusif au au détachement de salariés. Il conviendrait également, dans le cadre de l'action de lutte contre les pratiques de social et de concurrence déloyale, de refuser de voir les formulaires E101 et E102 s'appliquer à ces situations de détachement, qui ont un caractère fictif. Au-delà, il s'agit de s'assurer que les compagnies européennes exerçant une activité permanente en France versent les cotisations à l'URSSAF et aux régimes complémentaires de retraite. Monsieur le secrétaire d'État, quelles actions le Gouvernement compte-t-il prendre pour lutter contre ces pratiques de social et de concurrence déloyale courantes dans le secteur aérien, notamment de la part de certaines compagnies ? La parole est à M. le secrétaire secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, le Gouvernement est très attentif à la question du recours abusif par certaines compagnies aériennes au détachement des salariés pour exercer une activité pérenne sur le territoire national. Les autorités françaises ont mis en place un cadre juridique pour assujettir aux mêmes règles toutes les compagnies établies en France, dont les compagnies à bas coûts. Elles ont instauré la notion de « base d'exploitation », à savoir l'ensemble des locaux et infrastructures à partir desquels une compagnie exerce son activité de façon pérenne, là où les salariés prennent leur service et retournent à la fin de celui-ci. C'est la base d'exploitation qui définit le droit du travail applicable. C'est sur ce fondement

qui sera un élément supplémentaire pour mieux lutter contre les abus et détournements. En matière de protection sociale, les textes européens en vigueur, adoptés sur l'initiative de la France en 2012, prévoient que chaque personnel navigant est rattaché au système de sécurité sociale de l'État membre dans lequel se trouve sa base d'affectation. Dans le cadre de la révision engagée par la Commission des règlements portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, la France proposera des modifications des textes en vigueur précisant les modes d'organisation du travail adoptés par certaines compagnies. Plus généralement, la portée des formulaires attestant de la législation applicable en cas d'inexactitude, voire de fraude, devrait faire l'objet prochainement de précisions par la Cour de justice de l'Union européenne. Les autorités françaises soutiendront en outre une évolution des dispositions permettant la remise en cause des formulaires qui attestent d'une décision de législation de sécurité sociale erronée ou obtenue par fraude. La parole

Or, à l'heure actuelle, les solutions prétoriennes rendues en la matière se fondent sur le concept du trouble anormal causé, ce qui est loin d'être satisfaisant. Il incombe donc au propriétaire d'un monument historique de lourdes charges d'entretien de son bien immeuble, sans qu'il puisse bénéficier du contrôle de son image, alors que, paradoxalement, les créations architecturales récentes sont protégées par le droit d'auteur. Il semble à tout le moins logique que toute personne tirant des revenus commerciaux de prises de vues ou de l'image d'un monument historique contribue pour une part de ces revenus à l'entretien du monument concerné, sauf si le propriétaire y renonce explicitement.

Par ailleurs, et à titre de précision, j'insiste sur le fait que les dispositions concernant la liberté de panorama, votées à l'article 39 de la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, protègent protègent les reproductions et représentations d'oeuvres architecturales et de sculptures placées en permanence sur la voie publique faites par les particuliers pour leur usage personnel, notamment les réseaux sociaux Twitter, Facebook ou Instagram. Au vu de ces éléments, je vous remercie de nous faire part de votre position en la matière, madame la ministre, de même que des actions concrètes qui pourraient être engagées le cas échéant.

a été créée, par amendement parlementaire, pour cette catégorie spécifique de biens, dont la dimension symbolique, de par leur « lien exceptionnel avec l'histoire de la nation », justifie une protection toute particulière de leur image.

Cette liste a été soumise au ministre chargé des domaines, avant que les délimitations ne soient étudiées et soumises à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. Une liste de six domaines, dont le périmètre est clair et ne fait pas débat, lui a d'ores et déjà été présentée le 19 janvier dernier et elle a émis un avis favorable. Le décret correspondant vient d'être adressé au Conseil d'État. Les autres domaines nationaux, nécessitant des études plus importantes pour en arrêter le périmètre au vu de leur histoire, devront faire l'objet de décrets complémentaires. S'agissant des monuments historiques, la France compte environ 43 000 immeubles protégés à ce titre. Leur intérêt historique ou artistique est considérable, voire majeur, mais ils ne présentent pas, pour la plupart, la même dimension symbolique que les domaines nationaux.

Pour les monuments historiques dans leur ensemble, la jurisprudence de la Cour de cassation permet à un propriétaire d'obtenir une indemnisation dès lors que l'exploitation de la reproduction de son bien lui cause un trouble de jouissance anormal. Cette jurisprudence paraît suffisante, claire et appropriée. Comme vous l'indiquez vous-même, le droit à l'image sur les créations architecturales récentes est établi au bénéfice de son concepteur, comme c'est le cas pour toute oeuvre d'art ou de l'esprit. Les propriétaires, publics ou privés, des monuments historiques n'en sont pas les concepteurs, et ce droit ne saurait donc leur être transposé en l'état. Il nous semble donc préférable, dans l'immédiat, de nous en tenir à la mesure adoptée pour les domaines nationaux et d'en analyser la mise en oeuvre avant d'envisager toute généralisation à l'ensemble du patrimoine protégé. Enfin, je souhaite rappeler l'effort fait par ce gouvernement en direction des monuments historiques. Pour les seuls monuments historiques, la hausse des autorisations d'engagement a atteint 6 % en 2017, soit 355 millions d'euros. En moyenne annuelle,

diffusée par M6 les 17 août et 17 novembre derniers. Dans cette émission, qui était curieusement présentée comme un « documentaire-réalité

Beaucoup d'entre nous ont été choqués de la stigmatisation de populations en grande difficulté financière et sociale. Nous l'avons aussi été des clichés véhiculés par cette émission, dont l'alcoolisme ou le travail au noir. La FNARS, la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale, a appelé le Conseil supérieur de l'audiovisuel

». Bien qu'il ait déploré le choix du titre de l'émission, le CSA n'a, étonnamment, relevé aucun manquement de M6 à ses obligations

L'autorité indépendante a examiné cette émission. Vous l'avez rappelé, elle en a déploré le titre, à connotation péjorative et ne reflétant d'ailleurs pas la diversité des situations et des comportements des résidents du quartier de Saint-Leu à Amiens. a cependant estimé que M6 n'avait méconnu aucune des obligations que doit respecter une chaîne de télévision lorsqu'elle décide de mettre un programme à l'antenne En procédant ainsi, le CSA a exercé une mission que le législateur lui a confiée

On peut, bien sûr, sur un plan personnel, ne pas se retrouver dans la représentation donnée par cette émission. La réalité de la vie dans un quartier populaire est toujours bien plus complexe que la vision, forcément partielle, que peut en donner une caméra. Les médias assument naturellement une responsabilité éditoriale. Il appartient aussi au CSA, selon la loi, de contribuer « aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations dans le domaine de la communication audiovisuelle Mon souci constant, depuis un an, a été de renforcer l'action de l'instance de régulation sur ce sujet, et elle est désormais mieux armée. La loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a précisément renforcé sa mission sur ce point, en modifiant l'article 3-1. Désormais, la la loi prévoit explicitement que le CSA « veille à ce que la diversité de la société française soit représentée dans les programmes des services de communication audiovisuelle et que cette représentation soit exempte de préjugés

de décret relatif aux infirmiers anesthésistes diplômés d'État, les IADE, a été présenté en septembre 2016 ; il a reçu un avis favorable du Haut Conseil des professions paramédicales avant d'être transmis au Conseil d'État. Une concertation a ensuite été engagée entre la direction générale de l'offre de soins et les organisations syndicales représentatives, en vue de leur apporter un certain nombre d'avancées statutaires.

quasi-totalité du quinquennat. Avez-vous l'intention, madame la secrétaire d'État, de finaliser un accord qui prenne réellement en compte les attentes d'une profession, certes peu nombreuse, mais dont l'importance dans le fonctionnement des blocs opératoires est essentielle ?

Concernant ensuite la rémunération, la grille statutaire des infirmiers anesthésistes a évolué à deux reprises, en 2012 et en 2015. Dans la continuité du travail engagé sur l'évolution de l'exercice du métier, des négociations devant conduire à des revalorisations salariales ont été engagées. Un certain nombre de propositions ont été adressées aux organisations syndicales, d'abord dans le cadre d'un long processus de négociation avec le ministère de la santé, puis dernièrement dans une approche interministérielle, en association avec le ministère de la fonction publique. Ces propositions constituent un effort particulièrement important de la part du Gouvernement et démontrent l'attention spécifique accordée à la profession d'infirmier anesthésiste de bloc opératoire. Le résultat de ces négociations, qui sont toujours en cours, sera présenté

afin de faire face aux besoins des services d'urgence et d'obstétrique, avec un retentissement évident sur leur vie personnelle et familiale, sans que cela ne donne toujours lieu à des compensations adéquates. Actuellement,

d'oncologie. Les progrès de la recherche en cancérologie se sont accélérés ces dernières années. Ainsi, sur environ 355 000 nouveaux cas recensés chaque année dans notre pays, un cancer sur deux est guéri, notamment grâce aux meilleures performances de la recherche et aux différentes innovations thérapeutiques, qui contribuent également à améliorer la vie des patients atteints de cancer. Depuis plusieurs années, ces progrès ont abouti au développement de nouveaux médicaments, appelés thérapies ciblées, qui permettent de préserver au maximum les cellules saines environnant une tumeur. Plus récemment, les immunothérapies, traitements consistant à administrer des substances qui vont stimuler les défenses immunitaires de l'organisme, donnent des espoirs de guérison à des patients atteints de cancer jusqu'alors sans thérapies efficaces. Vraisemblablement, ce sont les associations de molécules, thérapies ciblées et immunothérapies, qui constitueront, dans un avenir proche, de nouvelles pistes pour combattre les tumeurs résistantes et offriront aux patients de nouvelles options thérapeutiques. Des réflexions sont en cours à l'échelle nationale sur le coût de ces traitements du cancer et sur les enjeux éthiques, qui ont fait l'objet de très nombreuses polémiques dans les médias. En conséquence, madame la secrétaire d'État, pouvez-vous indiquer au Sénat les actions que les pouvoirs publics, en particulier votre ministère, entendent mettre en place pour favoriser la recherche et l'innovation en oncologie ? Comment le coût de ces traitements et le développement de la recherche et de l'innovation ? Chacun sait en effet qu'une nouvelle molécule coûte extrêmement cher. Enfin, comment faire bénéficier plus rapidement les patients des résultats des essais cliniques,

ou à la combinaison de molécules thérapeutiques. C'est l'INCa, agence sous tutelle conjointe du ministère de la santé et du secrétariat d'État à la recherche, qui gère le PHRC-K. Par ailleurs, l'INCa, acteur national et international de premier plan, finance une douzaine d'appels à projets dédiés à divers aspects de la recherche en cancérologie, dont le développement de traitements innovants. L'institut est également en charge du suivi du troisième plan cancer et des actions en rapport avec la recherche et l'innovation dans ce domaine. Le ministère de la santé participe également activement au plan France médecine génomique 2025, piloté par dont une composante importante est la mise à disposition des techniques innovantes de séquençage à très haut débit pour le parcours de soins de patients souffrant de certains types de cancers, afin de leur offrir un traitement hautement adapté. Les deux premières plateformes seront ainsi financées en 2017 par le ministère de la santé et un projet pilote concernant l'utilisation du séquençage à très haut débit dans certains types de cancer est financé le PHRC-K. Le rapport d'étape du troisième plan Cancer, qui a été remis la semaine dernière au Président de la République, rappelle que la France entend poursuivre son effort de recherche, notamment fondamentale,

Monsieur le président, mon collègue Jérôme Bignon m'a demandé d'interpeller le Gouvernement sur les problèmes que nous rencontrons, d'une manière récurrente en France, en ce qui concerne le nombre de places disponibles pour l'accueil des enfants et adultes handicapés.

public- sécurité sociale ou département -, faute de réponses en France. Les établissements belges sont une alternative, mais ne constituent pas un recours pour tous ; ils sont principalement tournés vers les enfants atteints d'autisme, moins vers ceux qui présentent d'autres formes de handicap. Un programme visant à éviter ces départs a bien été lancé en 2015, avec un fonds d'amorçage de 15 millions d'euros. La première question que pose Jérôme Bignon concerne la pérennité de ce fonds et son inscription dans le temps pour la mise en oeuvre d'actions prioritaires.

sont dues à la situation des jeunes adultes handicapés, contraints de prolonger leur séjour en IME, faute de places dans des établissements adaptés à leur âge et à leur évolution. L'allongement de la vie pour nos concitoyens handicapés en est une raison.

Le 10 décembre dernier, un collectif départemental est né pour faire entendre la voix des familles exaspérées. La solution de l'inclusion scolaire, dont les moyens et les organisations sont d'ailleurs à revoir, s'avère inadaptée pour nombre d'enfants concernés, alors que des situations dramatiques ne peuvent être laissées sans recours. secrétaire d'État, quelles dispositions d'urgence l'État compte-t-il mettre en oeuvre pour permettre à ces enfants, adolescents et jeunes adultes d'intégrer, en temps, des établissements répondant à leur situation, les structures existantes pouvant dès maintenant les accueillir par simple extension de leur autorisation, comme le prévoit la réglementation actuelle ? La parole est à Mme la secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, vous m'interrogez sur les difficultés rencontrées par les parents d'enfants et d'adolescents en liste d'attente pour un institut médico-éducatif situé à Abbeville, dans la Somme.

désengorger l'IME, qui est géré par l'ADAPEI, un service d'éducation spéciale et de soins à domicile de dix places a été créé pour accompagner des enfants vivant avec des troubles du spectre autistique.

Je salue l'engagement résolu du Gouvernement face à cette problématique universelle, qui nécessite bien sûr une action coordonnée Une feuille de route a été annoncée au mois de novembre dernier afin d'intensifier la politique de maîtrise de l'antibiorésistance ; 330 millions d'euros vont être mobilisés sur cinq ans à cet effet. Cependant, en dépit de leur efficacité avérée au stade préclinique, l'utilisation des bactériophages, que je soutiens depuis des années, ne figure pas encore dans les mesures évoquées. Or, la phagothérapie, qui consiste à utiliser des qui consiste à utiliser des virus bactériophage pour traiter certaines infections d'origine bactérienne, constitue une voie très prometteuse, capable de répondre à des situations d'impasse thérapeutique. Cette solution

Madame la sénatrice, comme vous l'indiquez, l'utilisation de phages pour venir à bout d'infections bactériennes, en particulier à bactéries multirésistantes, est régulièrement évoquée.

En Europe, les bactériophages n'ont pour l'instant pas de statut spécifique, même si la définition du médicament est susceptible de leur être appliquée. En France, depuis 2013, l'essai clinique européen Phagoburn est en cours à l'hôpital d'instruction des armées Percy, à Clamart, avec pour objectif d'apporter des preuves sur l'efficacité de la phagothérapie. Cette étude est conduite en coopération avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des l'Institut suisse des produits thérapeutiques, Swissmedic, l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé belge, et l'Agence européenne des médicaments. À ce stade, il n'existe pas de recommandations européennes sur le développement des bactériophages. Néanmoins, Néanmoins, l'ANSM, par décision du 13 janvier 2016, a créé le comité scientifique temporaire Phagothérapie, dont vous avez parlé. Ce comité est chargé de donner un avis quant aux situations cliniques pouvant justifier un accès précoce aux bactériophages et aux prérequis nécessaires pour une mise à disposition précoce dans le cadre d'autorisations temporaires d'utilisation, les ATU, ou d'essais cliniques. Ce comité s'est réuni à plusieurs reprises au cours de l'année 2016. Un consensus s'est dégagé sur trois critères justifiant une situation de besoin, applicables à tout type d'infections pour un accès précoce aux bactériophages, à savoir un pronostic

du message à caractère sanitaire à destination des femmes enceintes qui, en application de l'article L. 3322-2 du code de la santé publique, doit figurer sur le conditionnement des boissons alcoolisées et qui prend, en pratique, la forme d'un pictogramme. Cette obligation résulte d'une initiative de la commission des affaires sociales du Sénat, qui s'est engagée de longue date pour la prévention des pathologies liées à l'alcool,

Dans le cadre de ses travaux de contrôle, notre commission a cependant constaté que la prévention de ce trouble devait urgemment être renforcée. Alors même qu'il est largement évitable, puisqu'il résulte principalement de la mauvaise information des femmes enceintes, le SAF continue en effet de constituer la première cause de handicap non génétique chez l'enfant. Dans les cas les plus graves, il peut entraîner la mort ; la plupart du temps, il est à l'origine de troubles neuro-développementaux divers, qui ont des effets pendant toute la vie. Face à ce fléau, la communauté scientifique comme la classe politique ont montré une mobilisation accrue au cours des dernières années, qui devrait porter ses fruits à moyen terme. Une action déterminante pourrait cependant être engagée dès aujourd'hui, par voie réglementaire, pour remédier à illisibilité du logo de prévention pour les femmes enceintes, caractère qui remet en cause sa pertinence. De très petite taille, il est en effet souvent à peine discernable, d'autant qu'il apparaît généralement en noir et blanc. Dans son rapport du 22 mars 2016, l'Académie de médecine relevait d'ailleurs que ce pictogramme est à totalement reconsidérer dans sa taille, son symbole, son positionnement et sa lisibilité ». Je souhaite savoir si le Gouvernement a d'ores et déjà engagé des travaux pour y remédier. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Les enquêtes périnatales l'ont montré, en 2010, 17 % des femmes enceintes déclaraient avoir consommé des boissons alcoolisées une fois par mois pendant la grossesse, et plus de 2 % d'entre elles en avaient consommé deux fois par mois ou plus, mettant ainsi en danger la vie de leur enfant. Depuis 2007, vous l'avez dit, toutes les unités de conditionnement des boissons alcoolisées doivent comporter soit un message sanitaire, soit un pictogramme, mais la lisibilité de ce pictogramme est clairement insuffisante. Nous savons que les fabricants favorisent l'harmonie du, au au détriment de la taille et de la lisibilité, c'est-à-dire des couleurs et du contraste utilisés. Ainsi, d'après l'enquête de la direction générale de la santé de 2012, un quart des buveuses déclarent ne même pas avoir remarqué ce pictogramme. Si, dix ans après sa mise en place, l'étiquetage d'informations sanitaires sur les bouteilles d'alcool

a décidé d'une mesure visant à améliorer la lisibilité et la visibilité du pictogramme, afin qu'il cesse d'être noyé dans le, au détriment de la santé publique. Des travaux interministériels vont s'engager

Dans l'Aisne, les jeunes souffrant de troubles psychiatriques peuvent être accompagnés par une unité de pédopsychiatrie pour adolescent en cas d'hospitalisation à temps plein. Pour les hospitalisations de jour ou le suivi externe, cet accompagnement est réalisé par une des équipes du centre psychothérapeutique pour adolescents. Selon son degré d'autonomie et d'avancement dans son parcours de soins, chaque jeune trouve une réponse adaptée à sa situation dans un délai raisonnable. Ces structures accueillent les patients jusqu'à l'âge À partir de 16 ans et 3 mois, les jeunes basculent vers la psychiatrie adulte. Alors que leurs maladies ne sont pas encore nécessairement installées et qu'ils apprennent à les appréhender, ils se trouvent en contact avec des patients adultes, à des stades différents de leurs maladies. Cette mixité pose problème tant dans la cohabitation des patients, néfaste pour les jeunes, que pour la prise en charge par les soignants, qui ne sont pas mesure d'adapter les actions de soin au public spécifique des jeunes. Partant de ce constat, les soignants de l'établissement de santé mentale départemental de l'Aisne proposent la mise en place, à titre expérimental, d'une structure spécifique, adaptée aux jeunes de 16 ans à 25 ans, pour assurer une continuité dans leur parcours de vie et de soins. En évitant les ruptures de prise en charge à un moment déterminant dans la construction personnelle, des hospitalisations graves et onéreuses pourraient ainsi être évitées. La structure envisagée devrait permettre d'accompagner le malade dans toutes les étapes, de la crise initiale à l'instauration d'un parcours de soin durable. Elle ferait le lien entre les nombreux partenaires que doit mobiliser un jeune adulte pour répondre à l'ensemble de ses problématiques. Dans l'Aisne, département largement touché par les suicides, par l'alcoolisme et les addictions, sous-doté en personnel médical, plus particulièrement en psychiatrie, une telle structure pourrait être un outil de santé publique pertinent. Il permettrait de corriger les inégalités de moyens constatées entre les établissements d'autres départements et ceux de l'Aisne, au bénéfice de patients déjà fragilisés par une situation sociale difficile et un personnel soignant en grande tension. C'est pourquoi j'ai souhaité appeler votre attention, madame la secrétaire d'État, sur ce projet d'expérimentation d'une nouvelle

Monsieur le sénateur, la question de l'extension de la psychiatrie infanto-juvénile jusqu'à l'âge de 18 ans a fait l'objet de préconisations dans le cadre de récents rapports-

Le Comité de pilotage de la psychiatrie, mis en place le 17 janvier 2017 sous la coprésidence du docteur Yvan Halimi et de la directrice générale de l'offre de soins, a identifié parmi ses thèmes de travail prioritaires la psychiatrie infanto-juvénile.

Sous l'impulsion constante du ministère des affaires sociales et de la santé, un maillage complet du territoire national en maisons des adolescents a été mis en place, pour accueillir les jeunes de 11 ans à 25 ans. La circulaire du Premier ministre du 28 novembre dernier relative à l'actualisation du cahier des charges des maisons des adolescents vise à renforcer davantage encore ce dispositif, qui a fait les preuves de son efficacité. Par ailleurs, de nombreux établissements ont mis en place des unités spécialisées pour adolescents et jeunes adultes qui permettent d'offrir une réponse au besoin d'hospitalisation dans un cadre moins stigmatisant qu'une unité d'hospitalisation traditionnelle et mieux adapté aux spécificités cliniques de l'entrée dans l'âge adulte. En 2014, on recensait 209 équipes spécialisées dans la prise en charge des adolescents. Le projet développé par l'établissement de santé mentale départemental de l'Aisne, sur lequel vous appelez l'attention de Marisol Touraine, vise à assurer aux jeunes de 16 ans à 25 ans présentant des troubles psychiques des parcours de santé et de vie de qualité, sécurisés et sans rupture. Mme la ministre demandera donc à l'agence régionale de santé des Hauts-de-France d'apprécier la faisabilité technique de cette expérimentation, qui paraît tout à fait intéressante, et d'étudier les modalités éventuelles d'un accompagnement financier sur des crédits du fonds d'intervention régional.

J'ai été récemment saisi du cas d'une personne confrontée à des conditions de vie très problématiques, en raison de l'isolement auquel elle est contrainte pour se protéger des radiations électromagnétiques artificielles. Il en résulte des conséquences très lourdes en termes de conditions de vie, d'accès à l'emploi, à la sociabilité et aux services essentiels. Cette situation risque Cette situation risque de surcroît d'être dégradée par l'autorisation accordée en 2015 à Orange de démanteler le parc de cabines téléphoniques. L'entreprise restait tenue de maintenir ce parc, en vertu du principe de service universel en matière d'accès au téléphone, lequel est désormais relativisé par le développement de la téléphonie mobile. Le retrait des dernières cabines téléphoniques en état de fonctionner risque de constituer une perte définitive, extrêmement préjudiciable, pour l'accès aux télécommunications. La personne ayant sollicité mon attention étant en effet contrainte de résider dans une habitation mobile, afin de rester éloignée des radiations, elle est dès lors privée de l'accès à la téléphonie fixe. L'exemple personnel sur lequel s'appuie ma question témoigne d'une situation très certainement partagée par plusieurs autres de nos concitoyens. Pour eux, la cabine téléphonique garantit un lien avec leurs proches et le monde extérieur. Je souhaite dès lors vous solliciter, madame la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, pour connaître les mesures qu'entend prendre le Gouvernement pour remédier à cette situation et aux conséquences négatives subies par les citoyens concernés. La parole

l'activité et l'égalité des chances économiques a retiré la composante « publiphonie » du périmètre du service universel des communications électroniques. Ce retrait a été largement avalisé par les élus locaux, en contrepartie de la relance des plans de couverture du territoire en services de téléphonie mobile. Cette évolution du périmètre du service universel, nécessaire et ayant recueilli l'assentiment des élus, s'est néanmoins accompagnée d'un certain nombre de précautions visant à garantir le caractère progressif et négocié du démantèlement des cabines. Orange s'est ainsi engagé, par lettre du 28 octobre 2015, à ne pas retirer de cabines dans des lieux qui ne seraient pas couverts par un service voix, à informer les maires au préalable et à organiser des réunions de concertation avec les élus concernés.

et l'hypersensibilité électromagnétique n'a pu être apportée jusqu'à présent ». Une expertise spécifique est en cours de réalisation au sein de la même agence. Le prérapport des travaux d'expertise a été mis en consultation publique du 28 juillet 2016 au 30 septembre 2016. Après examen des observations formulées lors de la consultation par les experts en charge des travaux, le rapport pourra être finalisé. Ce rapport et l'avis de l'ANSES devraient être publiés en 2017. Toutefois, les souffrances rapportées par les personnes indiquant être hypersensibles aux champs électromagnétiques ne peuvent être ignorées. C'est pourquoi une étude visant à mettre en oeuvre une prise en charge adaptée a été lancée en juillet 2012 par le service de pathologie professionnelle de l'hôpital Cochin de Paris. Il s'agit d'une étude pilote d'une durée de quatre ans, financée dans le cadre d'un programme hospitalier de recherche clinique. Les patients ont été reçus dans le centre de consultations de pathologies professionnelles et de l'environnement de leur région. Un suivi des symptômes des patients a été effectué durant un an. Le ministère des affaires sociales et de la santé s'appuiera, en 2017, sur les résultats de l'expertise de l'ANSES et sur ceux de l'étude coordonnée par l'hôpital Cochin pour établir, le cas échéant, des instructions concernant la prise en charge des personnes indiquant être hypersensibles aux champs électromagnétiques. Enfin, l'article 8 de la loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques, prévoit que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l'électro-hypersensibilité, rapport qui pourra faire état des orientations retenues sur une éventuelle prise en charge. Dans l'attente des conclusions du rapport scientifique de l'ANSES et de la publication des résultats de l'étude pilote, il nous semble prématuré d'introduire de nouvelles dispositions sur ce sujet.

la direction de l'AP-HP a décidé le départ des services de pointe de l'hôpital Jean-Verdier, notamment ceux de cancérologie et de chirurgie digestive. digestive. Un groupe de travail a par ailleurs été mis en place en vue de transférer, une fois encore, à l'hôpital Avicenne des services de Jean-Verdier que l'hépato-gastroentérologie, la réanimation, la radio interventionnelle, l'école d'infirmières, la maternité, la pédiatrie et la procréation médicale assistée- on est est presque essoufflé à la lecture de liste de tous ces départs programmés ! Cette décision est d'autant moins acceptable que l'on apprend, dans le même temps, que l'AP-HP se renseigne pour valoriser les terrains situés dans la zone ouest Jean-Verdier, où est implantée l'école d'infirmières, pour y réaliser une opération immobilière « juteuse », alors que cette parcelle pourrait accueillir des équipements médicaux de pointe. Par le démantèlement de ces services, c'est le droit à l'accès aux soins pour tous qui est menacé. L'hôpital Jean-Verdier doit rester un hôpital universitaire de proximité répondant aux besoins de la population. L'AP-HP doit pouvoir se développer autour de deux axes complémentaires, la médecine spécialisée de centre hospitalier universitaire et la médecine d'hôpital général de proximité,

Comme vous l'avez rappelé, il forme avec les CHU Avicenne et René-Muret le groupe hospitalier universitaire Paris-Seine-Saint-Denis depuis 2011. L'objectif du groupe hospitalier est de mutualiser des fonctions techniques et administratives entre les trois hôpitaux et de proposer des « parcours-patients » complets

et d'organiser les transformations de l'offre hospitalière en prise avec les besoins des habitants d'un territoire. Aussi, le groupe hospitalier universitaire Paris-Seine-Saint-Denis poursuit des réflexions sur l'organisation de l'offre de soins, notamment sur certaines disciplines de pointe et reconnues, aujourd'hui situées à Bondy, et dont la communauté médicale estime qu'elles pourraient bénéficier de synergies en se rapprochant des spécialités hospitalo-universitaires situées à Avicenne. Pour autant, si des réflexions médicales existent, elles ne préjugent pas des décisions qui seront ensuite arrêtées par la direction générale de l'AP-HP, qui devra s'assurer que ces orientations respectent effectivement l'impératif d'accès aux soins pour tous les habitants de ce territoire. Enfin, je saisis cette occasion pour vous rappeler combien l'AP-HP est précisément attachée à l'hôpital Jean-Verdier, dont les urgences adultes et pédiatriques, ainsi que l'unité médico-judiciaire, feront l'objet très prochainement d'une opération de modernisation de plus de 8 millions d'euros. Une structure ambulatoire innovante pourrait y voir le jour pour allier soins de proximité et excellence universitaire et mieux répondre aux besoins de la population, aujourd'hui confrontée à un fort déficit en consultations de médecine générale et de médecine spécialisée.

l'AP-HP a demandé à la communauté médicale non pas d'envisager son devenir, mais d'organiser le déplacement et le transfert de tous les services vers Avicenne.

La ligne est fréquentée par environ 600 personnes par jour. Celles-ci doivent aujourd'hui effectuer un trajet qui est relativement long, eu égard aux nombreux arrêts, et sur lequel on compte un nombre trop élevé de retards. Le projet de mettre fin à cette liaison directe et d'imposer un changement de train à Corbeil aurait immanquablement pour effet de dégrader les conditions dans lesquelles les usagers du Malesherbois effectuent leurs déplacements et d'en augmenter sensiblement la durée. De surcroît, il apparaît que 12 000 usagers environ prennent leur train dans les gares situées au sud de Corbeil seraient également touchés et verraient eux aussi leurs conditions de circulation dégradées. En outre, un tel dispositif se traduirait immanquablement par un report des circulations du train vers la voiture, nombre d'usagers du Malesherbois choisissant alors de se rendre à Étampes pour retrouver une liaison directe avec Paris. Cela n'irait pas dans le sens du respect de l'environnement, puisque cela accroîtrait la circulation et les besoins en stationnement. Un tel transfert serait également préjudiciable à tous ceux qui doivent se rendre, chaque jour, à Paris pour y travailler. Il apparaît donc souhaitable que

Je voudrais tout d'abord rappeler la constante préoccupation de M. le secrétaire d'État chargé des transports quant au renforcement et à la modernisation des réseaux existant de transports collectifs, ainsi qu'à l'amélioration des services. La qualité des transports du quotidien, pour tous, est essentielle. Le RER D a connu depuis le début des années deux mille une croissance annuelle de son trafic de 2,4 %, pour atteindre 615 000 voyageurs par jour. Cette croissance, comme les analyses le montrent, va se poursuivre. met évidemment à l'épreuve et l'infrastructure et l'organisation actuelle du service. La ponctualité du RER D ne s'élève aujourd'hui qu'à 85,5 %, et elle est même réduite à 64 % au sud de Corbeil-Essonnes. Entre 2010 et 2013, elle a perdu un point par an. Depuis 2014, les efforts de la SNCF et une réorganisation partielle du service ont permis de regagner quelques points, mais la hausse du trafic continue de peser sur la ponctualité, qui reste insatisfaisante. D'ici à 2025, la mise en oeuvre des schémas directeurs et le remplacement décidé de tous les anciens trains devraient améliorer considérablement la situation, mais, pour obtenir des résultats avant cette échéance, il est envisagé de modifier la structure de l'offre ferroviaire sur le RER D au sud. d'Île-de-France, qui est l'autorité organisatrice compétente, prévoit de modifier le plan de transport de la ligne. Le 11 janvier dernier, il a délibéré sur les évolutions à mettre en oeuvre, validant les grands principes du service annuel 2019.

de Goussainville à Châtelet, le soir ; deuxièmement, la complexité des circulations à Corbeil ; troisièmement, la saturation prévisible entre Melun et Paris le matin. Pour chacune de ces fragilités, des pistes d'action ont été étudiées. la simplification du noeud de Corbeil conduirait à réduire la longueur du RER D vers le sud et à envisager la suppression de la desserte directe de Malesherbes, qui ne fonctionne pas bien. Une correspondance robuste entre la branche de Malesherbes et le tronc principal du RER D serait alors organisée. Des avancées spécifiques seraient ainsi offertes aux passagers de cette branche grâce à de meilleures fréquences, notamment en soirée, et à la modernisation à venir du matériel roulant, comme vous l'avez indiqué, Ils bénéficieraient en outre de la régularité retrouvée sur le reste de la ligne D, et il en résulterait un temps de parcours vers Paris comparable à celui d'aujourd'hui, mais avec un confort sensiblement amélioré. Le secrétaire d'État aux transports a néanmoins pris note des réticences d'un certain nombre d'usagers sur cette nouvelle organisation. Il va donc demander au STIF d'examiner dans quelle mesure des trains directs pourraient être maintenus.

la possibilité de maintenir une ligne directe. Je puis vous dire que, avec les élus concernés, je vais de mon côté prendre contact avec la SNCF et le STIF

de plan État-région 2015-2020 préconise la mise en oeuvre de dispositifs d'amélioration de la desserte du littoral, dont la sécurisation de la RN 248, à hauteur de la commune.

La priorité d'aménagement est la mise en deux fois deux voies de la RN 11 au droit du contournement de Mauzé-sur-le-Mignon, ainsi que la sécurisation de la RN 248 par l'aménagement du carrefour de Frontenay-Rohan-Rohan, d'un coût total de l'ordre de 26 millions d'euros. Sur la période 2015-2020, le montant des premiers aménagements et engagements est de l'ordre de 16 millions d'euros. Cette opération d'aménagement routier a été retenue dans le cadre du volet mobilité multimodale du

Je vous serai reconnaissant de bien vouloir nous indiquer dans quel délai nous pouvons espérer la mobilisation des premiers crédits et nous communiquer le calendrier des travaux de sécurisation de ces carrefours, laquelle devrait déjà être achevée. Je vous remercie des éléments que vous serez en mesure de nous fournir. La parole

Je tiens à vous assurer que l'État a pleinement conscience de l'importance des enjeux de sécurité sur cet itinéraire, qui supporte un trafic de l'ordre de 7 500 véhicules par jour, dont 13 % de poids lourds. Comme vous le soulignez, une enveloppe de 16 millions d'euros est inscrite au contrat de plan État-région 2015-2020, afin d'améliorer la desserte du littoral depuis l'A 10. La sécurisation de la RN 248, par l'aménagement de ses carrefours, est notamment citée. Deux carrefours avec le réseau secondaire départemental sont identifiés dans le cadre de cet aménagement : celui avec la RD 118, dit carrefour du silo, et celui avec la RD 102. Ceux-ci, qui sont situés sur la commune de Frontenay-Rohan-Rohan, sont très rapprochés, à moins de 1,5 kilomètre. Alain Vidalies est conscient de la nécessité d'un aménagement améliorant la gestion des flux des réseaux secondaires, en organisant l'échange en un seul point avec la RN 248 par un carrefour dénivelé. Toutefois, l'important programme d'opérations engagé, tant en travaux qu'en études par les services de l'État en région, ne permet pas de commencer cette opération dès 2017 au vu des disponibilités budgétaires. Les études d'opportunité visant à identifier le meilleur parti d'aménagement seront donc lancées à partir de 2018. Une fois celui-ci approuvé, les études techniques et environnementales seront conduites et les acquisitions foncières réalisées afin de pouvoir engager les travaux tels qu'ils sont prévus par l'actuel contrat de plan.

ceux-ci devaient débuter en janvier sur le tronçon Carcassonne-Limoux, la direction régionale de SNCF Réseau aurait planifié la fermeture du segment Limoux-Quillan pour la fin de l'année 2017. Je tiens donc à rappeler ici que, dans le cadre du contrat de plan État-région, ces deux partenaires et la SNCF se sont engagés dans le processus de rénovation et d'exploitation sur la totalité de la ligne Carcassonne-Quillan. J'y insiste : la totalité

Une telle annonce est inacceptable, d'autant que cette ligne connaît depuis plusieurs années une fréquentation en hausse. Permettez-moi de souligner, une fois encore, l'importance de cette infrastructure pour le développement économique de ces territoires. Les projets de fret sur cette ligne sont nombreux, mais ils ne se concrétisent pas, faute d'opérabilité de cet outil. Je ferai la même remarque concernant les projets touristiques.

la ligne doit rester en totalité dans le périmètre de l'État ; la continuité des circulations ferroviaires doit pouvoir être assurée, et il convient donc d'effectuer les travaux de maintenance et d'entretien nécessaires ; le tronçon Limoux-Quillan devra, pour sa régénération, être inscrit au contrat de plan État-région de 2021. Je crois d'ores et déjà pouvoir assurer que le conseil régional s'engagera pour cette deuxième tranche de travaux.

L'État et la région ont souhaité inscrire dans le CPER 2015-2020 une enveloppe de 11 millions d'euros. D'après les études, ce montant permet de traiter la section entre Carcassonne et Limoux, où circulent le plus grand nombre de trains. C'est donc un engagement fort en faveur de cette ligne et de la haute vallée de l'Aude qui a été pris dans le cadre du CPER. L'ensemble des partenaires, dont l'État, ont mobilisé en 2016 les crédits nécessaires au lancement des travaux sur cette section. La première phase s'achèvera en mars 2017, tandis que la seconde sera réalisée au premier trimestre 2018. La rénovation de l'ensemble de la voie ainsi que de six ouvrages d'art sur fonds propres de SNCF Réseau permettra d'assurer la pérennité des circulations pour une quinzaine d'années. S'agissant de la section Limoux-Quillan, dont vous appelez la rénovation de vos voeux, de vos voeux, les travaux correspondants représenteraient, pour cet itinéraire de 30 kilomètres, un investissement de l'ordre de 40 millions d'euros, qui n'est pas financé à ce jour. De façon plus générale, l'avenir de la ligne Carcassonne-Quillan, ligne de desserte fine du territoire, doit être envisagé à l'échelle régionale afin d'identifier les réponses les plus pertinentes à apporter en termes de mobilité durable, en fonction des caractéristiques des territoires. L'initiative du nouvel exécutif de la région Occitanie d'organiser des états généraux du rail et de l'intermodalité, qui a été un moment fort de concertation entre tous les citoyens et les acteurs locaux, va dans ce sens. Leur restitution en décembre dernier a mis en exergue la nécessité de sauvegarder la ligne Carcassonne-Quillan avec cinq autres lignes régionales identifiées comme prioritaires. Le soutien financier de l'État aux lignes de desserte fine du territoire s'inscrit dans le cadre des contrats de plan État-région, comme c'est le cas pour la section Carcassonne-Limoux. Dans ces conditions, les investissements en faveur de la section Limoux-Quillan devront donc soit relever d'une intervention des collectivités territoriales, en fonction de leurs priorités au au niveau régional, soit être abordés dans le cadre de la prochaine révision du contrat de plan.

de la biodiversité sur les actions conduites par la France pour réviser les dispositions ayant trait à la protection des loups dans la convention de Berne du 19 septembre 1979, laquelle est en application depuis le 1 juin 1982. S'il est vrai qu'en 1979 le nombre de loups était très limité, force est de constater qu'il n'en va plus de même puisqu'on estime désormais à environ 500 le nombre de loups sur le sol français. Au départ signalée uniquement dans les Alpes du Sud, la présence du loup est désormais avérée dans tous les massifs français de l'est de la France, jusqu'en Lorraine. Cette prolifération est également rapide

traumatismes, mécontentements et fortes inquiétudes des éleveurs d'ovins, de chèvres et même de jeunes bovins, qui doivent faire face aux attaques répétées de leurs troupeaux par les loups. À quand les humains ? Veut-on complètement décourager nos éleveurs d'ovins, alors même qu'ils doivent déjà faire face à de nombreuses autres contraintes ? Va-t-on encore longtemps considérer le loup comme une espèce protégée, laissant les éleveurs face à d'innombrables contraintes pour protéger leurs cheptels ? ? Alors que l'on attend à juste titre des éleveurs qu'ils aient le souci du bien-être animal, va-t-on encore tolérer pendant longtemps que les loups déchiquètent de façon horrible plus de 9 000 ovins et caprins chaque année,

Enfin, que comptez-vous faire pour les éleveurs, aujourd'hui pris en tenaille entre l'obligation de protéger leurs troupeaux des loups avec des chiens patous et les ennuis, voire les procès, que les agressions causées par ces chiens à des randonneurs peuvent leur valoir ?

Au vu de tels chiffres, qui peut croire que le loup soit une espèce en voie de disparition ? C'est pourquoi, madame la secrétaire d'État, je souhaite que vous indiquiez à la représentation nationale si le Gouvernement a fait une demande de révision de la convention de Berne au sujet du loup. Dans

Le loup est une espèce protégée au titre de la convention de Berne et de la directive européenne habitats-faune-flore. La France se doit de respecter strictement ses engagements internationaux et donc d'assurer la protection et le bon état de conservation d'une population estimée aujourd'hui à 300 loups sur l'ensemble du territoire.

sur le long terme, partagée par tout le monde. C'est pourquoi j'ai lancé le 7 juillet dernier une démarche d'évaluation prospective du loup en France à l'horizon 2025-2030. Elle comprend deux volets. la réalisation de deux expertises collectives pour disposer des données scientifiques qui doivent rester la base de notre action : l'une sur la biologie de l'espèce et sur sa répartition sur le territoire ; l'autre sur les aspects sociologiques et les relations entre l'homme et le loup, car on sait que cet animal s'adapte et réagit aux mesures aux mesures mises en place face à lui. Ensuite, il y a l'élaboration d'une stratégie à l'horizon 2025-2030, en concertation avec tous les acteurs concernés. Bien évidemment, les éleveurs et les organisations agricoles sont autour de la table. J'ai la conviction que la politique a un rôle à jouer sur la question du loup, comme pour d'autres espèces, et peut-être plus encore compte tenu du symbole que représente le loup. Il faut bien avoir à l'esprit que, depuis près de cent ans, les éleveurs ont vécu sans le loup,

Dans le récent rapport d'information parlementaire consacré à la mise en application de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, il a été rappelé le rôle déterminant de l'hydroélectricité dans le mix énergétique français et dans la transition énergétique à venir. Ce rôle est d'ailleurs confirmé par la programmation pluriannuelle de l'énergie, récemment publiée, et qui consacre une place centrale à l'hydroélectricité comme complément idéal des productions éoliennes et solaires, et appelle de ses voeux des développements nouveaux de cette énergie. La loi a introduit la possibilité pour l'État de prolonger des concessions hydroélectriques pour y réaliser des investissements. Il semble que cette option soit retenue pour les concessions de la vallée du Rhône. Or des projets s'inscrivant les objectifs de la loi de transition énergétique existent sur les vallées d'importance nationale du Lot et de la Truyère. Ces projets pourraient être lancés rapidement dans le cadre d'une prolongation. Ils auraient un impact très positif sur le développement de nos territoires ruraux, en termes tant d'emplois que de ressources nouvelles pour nos collectivités. Alors que nos territoires ont tant besoin d'investissements et que notre pays doit relever le défi de la transition énergétique, pourriez-vous nous préciser les intentions du Gouvernement s'agissant de la prorogation des concessions du Lot et de la Truyère ? secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte consolide le régime des concessions hydroélectriques et garantit le respect des enjeux de service public de l'hydroélectricité française : accélération du développement des énergies renouvelables ; sécurité d'approvisionnement en électricité ; sûreté des barrages ; sécurité des personnes ; contribution à la continuité écologique des cours d'eau et, enfin, ancrage territorial des concessions, qui contribuent au développement économique local, avec le maintien des compétences et des emplois dans les barrages et les usines. Le Gouvernement défend une mise en oeuvre équilibrée de la loi grâce à différents outils : le regroupement des concessions, la prolongation des concessions en contrepartie d'investissements et la possibilité de constituer des sociétés d'économie mixte lors du renouvellement des concessions. Dans ce cadre, le Gouvernement soutient la réalisation de nouveaux investissements pour le développement de l'hydroélectricité. Certains pourraient être réalisés dans le cadre d'une prolongation de concession existante, qui devra alors respecter qui devra alors respecter les droits français et européen applicables aux contrats de concession. Ce dossier fait actuellement l'objet d'échanges avec la Commission européenne, dans le cadre de la procédure ouverte par la mise en demeure adressée en octobre 2015 à la France. Le traitement des concessions hydroélectriques dans la vallée du Lot et de la Truyère s'inscrira dans la réponse globale équilibrée que la ministre recherche avec la Commission européenne. En tout état de cause, le régime concessif des installations hydroélectriques permet un contrôle public fort, au travers de la réglementation et des contrats signés entre l'État et le concessionnaire. Il permettra donc d'assurer la réalisation des investissements souhaités

ministre de l'intérieur. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, ma question porte sur l'avancement du projet de rénovation du commissariat de police d'Épernay, dont l'état de conservation ne permet pas aux fonctionnaires de travailler et de recevoir les usagers dans des conditions adéquates.

Même si des travaux d'urgence ont été effectués, ceux-ci ne suffisent pas. Ce dossier constituait, il y a quelques mois, l'un des sujets prioritaires de la zone du secrétariat général pour l'administration de la police de Metz. Il a été rejoint aujourd'hui par le commissariat de Reims, qui est aussi particulièrement dégradé. Je tiens à vous rappeler les propos de votre collègue Hélène Conway-Mouret, le 19 novembre 2013, en réponse à la même question : « En ce qui concerne le commissariat d'Épernay, ses locaux sont effectivement vétustes et inadaptés aux besoins des services. [ Si les contraintes budgétaires extrêmement fortes n'ont malheureusement pas permis l'inscription de cette opération dans la programmation budgétaire triennale 2013-2015, vous pouvez être assurée que ce dossier continuera de faire l'objet de toute l'attention du ministre et de ses services, qui sont parfaitement conscients de son importance, tant pour les habitants et leurs élus que pour les fonctionnaires de police. » Or, depuis, rien n'a été entrepris le Gouvernement s'était déjà engagé, fin décembre 2012, à traiter ce dossier avec la plus grande attention et à examiner sa faisabilité dans le cadre de la prochaine programmation triennale, programmation aujourd'hui échue Le 26 octobre dernier, le Premier ministre a fait part « d'une enveloppe globale de 250 millions d'euros et d'une enveloppe supplémentaire afin d'assurer l'entretien du parc immobilier et les travaux de maintenance les plus urgents dans les commissariats de police et les casernes de gendarmerie la secrétaire d'État, que les crédits ne sont pas encore arrivés dans la Marne ! Au regard des différents engagements de vos gouvernements, le commissariat d'Épernay doit faire l'objet d'une requalification complète des locaux.

secrétaire d'État. Madame la sénatrice, les conditions de travail des policiers sont un sujet essentiel. Aux policiers, aux citoyens et aux victimes, l'État se doit d'offrir des commissariats à la hauteur des exigences d'un service public moderne et respectueux de ses agents et de leur engagement quotidien. C'est pour toutes ces raisons que les crédits d'équipement et d'investissement des forces de l'ordre sont en hausse depuis le début du quinquennat. Toutefois, les besoins sont considérables et de trop nombreux commissariats de police sont dans un état indiscutablement médiocre, voire inadapté ou vétuste. C'est la raison pour laquelle le ministre de l'intérieur a lancé, fin octobre, un important plan sécurité publique, qui représente une enveloppe globale de 250 millions d'euros. Il prévoit en particulier une enveloppe budgétaire de 16 millions d'euros dédiée à l'immobilier pour pallier les problèmes les plus urgents de vétusté et d'inadaptation de certains commissariats. Ces crédits ont été délégués dès le 4 novembre directement aux services territoriaux de police. S'agissant du commissariat d'Épernay, ses locaux sont indiscutablement vétustes et inadaptés aux besoins. Des travaux de réhabilitation d'urgence et de rénovation sont donc régulièrement réalisés, et ce depuis plusieurs années. En 2015 et 2016, par exemple, l'accueil a été rénové et des travaux de sécurisation du site ont été effectués. Par ailleurs, grâce aux crédits exceptionnels du plan sécurité publique, des travaux ont été réalisés en urgence au commissariat d'Épernay- équipements de sécurité incendie et réfection de la tuyauterie sur le circuit de chauffage. D'autres travaux sont encore nécessaires. À plus long terme, il faudra- vous avez raison -aller bien au-delà. Plusieurs hypothèses de relogement du commissariat ont été examinées ou évoquées au cours de ces dernières années construction neuve sur le site actuel, construction neuve sur un autre terrain, extension-réhabilitation du bâtiment existant. Cette dernière option semble techniquement la plus fiable et les services locaux ont déjà travaillé en 2014 et 2015 sur le programme technique détaillé. dans le contexte budgétaire contraint que vous connaissez, cette opération, qui se monterait en études et en travaux à plus de 6 millions d'euros, n'a pas encore pu être programmée.